Depuis, cette idée a circulé, elle a convaincu, au delà de notre groupe, ce dont nous nous réjouissons. Aussi, nous avons l’occasion de faire adopter ici une véritable taxation des comportements strictement spéculatifs pour, sinon les dissuader, du moins en retirer une manne financière, estimée au minimum à 1,5 milliard À peu de chose près, voter en faveur de cet amendement justifierait de ne pas augmenter les taxes sur l’électricité ou de ne pas sous valoriser les pensions de retraite, ou encore de ne pas faire travailler gratuitement les salariés et fonctionnaires de ce pays : sur ce dernier point, il y a eu un rétropédalage, c’est le moins qu’on puisse dire

Du point de vue fiscal, elle vise à mieux prendre en compte l’ampleur de ce phénomène. La part des rachats dans le montant total des sommes distribuées par les entreprises du CAC 40 a ainsi presque doublé en sept ans, passant de 8 % en 2017 à 15 % en 2023. Le montant annuel des rachats a par ailleurs été multiplié par 2,5 sur cette période. Une telle opération, qui gonfle artificiellement le montant des actions, est aujourd’hui favorisée par une absence de traitement particulier au sein de la fiscalité française.

artificiellement la valeur des actions restantes, ce qui accroît mécaniquement les bénéfices et, en conséquence, les dividendes versés. Voilà l’illustration parfaite de la financiarisation de notre économie et de ses dérives. Un tel dispositif privilégie privilégie exclusivement les actionnaires, sans apporter de bénéfices réels à l’investissement productif ni à l’emploi. Ces pratiques, qui n’ont pas de justification économique, méritent d’être beaucoup plus fortement encadrées, voire dissuadées, par une taxe additionnelle. Rappelons qu’en France,

à leur valeur réelle à 4 % permettrait de générer des recettes fiscales importantes sans pour autant pénaliser les investissements productifs ni affaiblir la compétitivité des entreprises. Certes, j’ai bien entendu l’argument fondé sur le régime mère filles,

La logique voudrait que l’on modifie globalement l’assiette en retenant la valeur de rachat des titres annulés. Si le Gouvernement n’a pas souhaité retenir cette solution, c’est parce que, comme cela a été dit, il existe de forts risques qu’elle soit

Je veux qu’à cet instant chacun se souvienne du sort réservé à la taxe instituée en 2012. Après sa censure

laisser subsister que la valeur de rachat des titres annulés et à adapter le taux pour le faire correspondre à cette nouvelle assiette.

: La parole est à Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Corinne Bourcier vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre

et d’éviter toute distorsion dans la concurrence entre celles ayant réalisé les opérations avant la date d’application de la loi et

merci. capital les opérations résultant de l’annulation de titres rachetés soit aux salariés qui les détiennent dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié, soit à un fonds commun de placement à travers lesquels les salariés les détiennent indirectement, soit à une entité les ayant acquis dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir leur liquidité.

vise à exclure du champ de la taxe les organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés et de sociétés de capital risque. Quel est l’avis de la commission

Je le dis sans équivoque, et j’espère que le message sera bien entendu par ses destinataires : ce ne sont pas les banques qui font la loi dans ce pays ! En France, cinq grandes banques sont actuellement poursuivies par l’administration fiscale et par le parquet national financier (PNF) pour de telles manipulations, et le fisc a déjà notifié 2,5 milliards d’euros de redressement aux établissements incriminés. Ces derniers auront eu recours à toutes les manœuvres dilatoires possibles et imaginables : dénégation sur l’abus de droit

pensant être protégés par la complexité ou l’opacité des montages qu’ils mettent en œuvre. Je le dis clairement : la complexité n’implique pas l’impunité.

Cette notion de « bénéficiaires effectifs » – j’y insiste – est entrée dans le droit en 2001 aux Pays Bas. Nous sommes loin d’être les pionniers en Europe. Au Danemark, son inscription a permis l’augmentation de 130 % des montants de retenue à la source depuis 2015 ; cela nous donne des raisons d’espérer. Et, dans ces pays, les banques n’ont pas perdu en compétitivité, sauf, évidemment, sur le marché des montages financiers frauduleux. De même, l’attractivité de la place de Paris ne sera pas remise en cause, malgré ce que de nombreux acteurs nous prédisent. Ensuite, l’amendement tend à redonner sa vigueur au dispositif anti abus qui a été adopté, ici, au Sénat, et qui a malheureusement été rendu inopérant lors de la navette parlementaire. Nous y intégrons des opérations complexes réalisées des marchés réglementés ou par des produits dérivés ; il ne serait pas sérieux de les exclure si l’on cherche véritablement à mettre fin aux CumCum.

C’est ce qu’il faut faire. C’est d’ailleurs devenu une évidence : tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale aux CumCum le disent. Tous les pays qui ont lutté efficacement contre les pratiques en question

du sous amendement créerait un trou béant dans la raquette. On sait aujourd’hui que la grande majorité des montages CumCum ont lieu des marchés réglementés. Et sous prétexte que ces opérations seraient les plus opaques,

C’est précisément parce que le destinataire est incertain que la retenue à la source doit s’appliquer, au moins par défaut. C’est ce que font, notamment, les États Unis. Que je sache, ce ne sont pas tout à fait les ennemis de la finance, et ils ne sont pas non plus réputés pour vouloir asphyxier le système bancaire Il ne me paraît pas sérieusement envisageable d’exclure les transactions dans lesquelles la banque peut démontrer qu’elle n’a pas perçu elle même le dividende. Les banques savent détacher le titre chez un tiers, afin de clamer qu’elles n’ont jamais reçu le dividende à taxer. En excluant ces transactions, nous créerions de nouveau une prime, pour ne pas dire une récompense, à l’opacité en ne couvrant pas une pratique déjà avérée. Monsieur le ministre, je constate avec étonnement

Le Gouvernement souhaite t il s’engager résolument ou non contre la fraude fiscale à grande échelle de certains établissements financiers ? C’est la question qui nous est posée. Vous connaissez la réponse que nous y apportons.

l’avis du Gouvernement

Monsieur le ministre,

à compter du 31 décembre 2024 pour les seules entreprises ayant subi des déficits excédant ce plafond au titre des deux derniers exercices 2023 et 2024. Autrement dit, il s’agit

L’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Même si cette taxe finance notamment l’aide publique au développement, une telle augmentation pourrait contribuer utilement au financement du rehaussement de l’ambition écologique mondiale. Le récent échec de la COP16 sur la biodiversité, délocalisée de Colombie à Rome dans l’espoir que ce nouveau tour de négociation débouche sur un accord sur le financement, démontre la nécessité de taxer la spéculation.

Cet amendement vise à augmenter les recettes assises sur les transactions financières et à élargir l’assiette de la TTF aux transactions intrajournalières. Cette mesure est doublement pertinente : le risque de contournement apparaît modéré et le ciblage des opérations intrajournalières vise les activités les plus spéculatives.

et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement au travers du fonds de solidarité sur le développement, il est possible de garantir une contribution équitable du secteur financier, tout en refusant

Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, la France fait face à des défis majeurs sur la scène internationale, en particulier en Afrique. Les récents événements au Tchad et au Sénégal, symboles d’une érosion de notre influence, rappellent l’urgence de redoubler d’efforts plutôt que de céder à la tentation du repli. Réduire notre aide au développement en ces temps troublés serait non seulement un renoncement, mais aussi un message de fragilité adressé à ceux qui aspirent à voir la France reculer dans le concert des nations. L’aide au développement est bien plus qu’un moyen financier. Elle porte en elle une promesse de solidarité, une capacité à réparer les fractures complexes et à offrir un avenir partagé. Il est impératif de redéfinir notre relation avec l’Afrique, en rompant avec les perceptions réductrices

permettront de redorer notre image, de renforcer nos alliances et de bâtir une relation fondée sur la coopération, l’échange et le respect mutuel. C’est par cette ambition empreinte de fraternité et d’humanisme que la France peut continuer à jouer un rôle moteur sur la scène internationale. La TTF permet de défendre ces principes et de les réaffirmer sur la scène internationale.

l’avis du Gouvernement ?

monsieur le ministre

cet amendement, notre collègue Annick Billon propose une solution de financement durable pour les littoraux subissant l’érosion côtière.

locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être versé au fonds érosion côtière,

cet amendement, mon collègue Jacques Fernique propose de créer une taxe pénalisant les deux roues et trois roues motorisés les plus bruyants. Alors qu’ils ne représentent que 2 % du transport routier de voyageurs, ces véhicules contribuent de manière disproportionnée à la pollution sonore, enjeu majeur de santé publique.

Ces conflits modernes mettent d’ailleurs en lumière le double standard et le « deux poids, deux mesures » dans l’application du droit international. Nous sommes convaincus que l’arme la plus efficace pour construire la paix et sauver notre humanité ne doit être que celle du droit. Le bilan de l’acharnement barbare à Gaza est à rappeler sans cesse : plus de 44 000 morts, dont 70 % de femmes et d’enfants, d’innombrables disparus, présumés morts sous les décombres, l’exode massif de populations à la recherche éperdue d’un refuge qui n’existe pas. Dans un monde ordonné et stable, le droit ne saurait être une simple superstructure accessoire. Notre groupe n’a d’autres repères dans le monde que le droit international incarné par les Nations unies, quand bien même l’un et l’autre sont perfectibles.

il nous est apparu comme un minimum de rendre automatique une hausse des tarifs douaniers pour tout pays ne respectant pas les recommandations émises par une résolution en émanant. Aujourd’hui, les deux pays ne respectant pas ce type de résolution sont la Russie et Israël. Si, dans le premier cas, nous n’avons pas tremblé pour sanctionner l’appareil productif de la Russie de Poutine, notre pays reste aphone concernant Israël.

anciennement classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans le nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et proroge le dispositif d’exonération fiscale et sociale dans les bassins d’emploi à redynamiser

Merci

dérogation à la date limite de délibération, afin de permettre aux collectivités d’instaurer, avec un effet pour les impositions au titre de 2025, certains dispositifs d’exonération s’appliquant en FRR : exonération facultative temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements qui sont acquis, puis améliorés, au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en vue de leur location ; exonération facultative temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux. tend également à proroger jusqu’au 31 mai 2025 l’effet des délibérations des conseils départementaux, pris avant le 15 avril 2024, instaurant l’abattement de DMTO applicables dans les ZRR. à renforcer les clauses anti abus du régime zoné des FRR prévues pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux délocalisations et aux transferts d’entreprises. À ce titre, il est proposé de décompter le délai de cinq ans de la clause anti délocalisation à partir, non pas de l’année où l’entreprise bénéficie pour la première fois de l’exonération, mais de l’année où elle en bénéficie pour la dernière fois.

sur 564 étaient classées en ZRR. Or le nouveau mode de calcul a sorti 89 communes du dispositif. Ces dernières ont notamment été victimes du calcul du revenu moyen disponible, désormais

inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine.

de type rural si plus de 60 % de sa population vit en zone rurale, et de type rural autonome si moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.

premier lieu, le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui sert de base à ces critères, n’est pas encore disponible dans ces territoires. Sa mise en œuvre a été reportée à 2028 pour les outre mer et à 2030 pour Mayotte, ce qui bloque la mise en œuvre de ce dispositif.

Cet amendement tend non pas à remettre en cause les objectifs environnementaux de long terme, mais à adapter le dispositif aux réalités locales. Il est essentiel pour permettre aux territoires ultramarins de bénéficier pleinement de cette aide et pour soutenir la réhabilitation de leur parc social dès maintenant. Je vous invite donc à voter en faveur de cet amendement pour défendre un habitat digne et accessible dans l’ensemble de nos territoires ultramarins. L’amendement

Canévet tend à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, certains dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivent à échéance en fin d’année.